monsieur le président La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2020 Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'ensemble des salles de réunion et des circulations du Sénat. Il vous est donc demandé de bien vouloir en porter un dans l'hémicycle.

les mesures de relance. Je considère que le plan de soutien du Gouvernement dans ce PLFR aurait dû être amplifié sans attendre la mise en oeuvre d'un plan de relance à la rentrée-

que les ménages et les entreprises ont besoin dès à présent de visibilité pour prendre leurs décisions en matière d'investissement et de consommation. Pour autant, au-delà de ce sujet- nous avons pris date sur la relance -et dans le même esprit que celui qui nous a guidés lors du vote des PLFR 1 et 2, le Sénat a, en conscience et responsabilité, voté, dès la première lecture, les mesures de soutien du Gouvernement et le renforcement des dispositifs qui ont démontré leur utilité : prêts garantis par l'État, par l'État, fonds de solidarité, mais aussi compensation des pertes des collectivités territoriales. Certes, nous souhaitions des améliorations de tel ou tel dispositif, mais, sur le fond, nous étions d'accord. Laurent

la compensation des pertes de recettes des collectivités territoriales grâce aux apports du Sénat. Tout d'abord, s'agissant des départements, est conservée la clause « de retour à meilleure fortune »- on peut la qualifier ainsi

dans cette assemblée que les Franciliens voyagent dans de bonnes conditions et que le matériel ne doit pas être renouvelé. Si l'absence de compensation ou l'insuffisance de compensation par l'État devait entraîner l'arrêt des commandes, cela aurait bien sûr des conséquences pour les Franciliens, qui continueraient de voyager dans de mauvaises conditions, mais également pour l'emploi, car les commandes de matériels sont source d'emplois, y compris dans nos régions. Deuxièmement, afin de renforcer le soutien aux entreprises les plus fragilisées- c'était important pour le Sénat le dispositif de remises de dettes partielles prévu à l'article 18 a été étendu à l'ensemble des entreprises de moins de 250 salariés qui auraient perdu plus de 50 % de leur chiffre d'affaires.

La CMP a également conservé, bien évidemment, les importantes hausses de crédits votées par le Sénat, sur l'initiative du Gouvernement. Je pense aux crédits supplémentaires pour le renouvellement du parc automobile de la police et de la gendarmerie nationales, à hauteur de 60 millions d'euros- sujet cher à notre rapporteur spécial Philippe Dominati. Je pense également à l'augmentation des moyens des Crous, pour 50 millions d'euros,

Concernant la prime à l'embauche, nous nous félicitons que des crédits aient été prévus à cet effet. Le Sénat avait voté l'enveloppe que j'avais proposée, qui était un peu plus importante. Le texte de la CMP reprend les montants du Gouvernement, qui ne sont pas si éloignés. Certes,

J'estime essentiel de soutenir plus spécifiquement les PME dans leurs recrutements dès lors qu'il s'agit de jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs généraux, mesdames, messieurs les sénateurs,

Je pense notamment au financement du chômage partiel ou du fonds de solidarité. Je pense aussi à tous les dispositifs que nous avons mis en place et qui permettront d'amplifier les efforts en direction du secteur industriel ou de garantir l'accompagnement de nos compatriotes les plus fragilisés.

à la moyenne des recettes de la période 2017-2019, un traitement particulier étant prévu pour les outre-mer afin de prendre en compte leurs spécificités, notamment le droit d'octroi ou la taxe spéciale sur la consommation.

Le dispositif qui a été adopté permet ainsi d'exonérer l'ensemble des TPE ayant fait l'objet d'une décision de fermeture administrative, ainsi que, pour quatre mois, les TPE et les PME des secteurs les plus touchés- on pense immédiatement aux cafés, aux hôtels ou aux restaurants, mais pas seulement : le sport, la culture, l'événementiel sont concernés. Nous avions prévu un dispositif d'exonération partielle et au cas par cas pour les entreprises de moins de 50 salariés ; vous avez fait le choix, mesdames, messieurs les sénateurs, retenu en commission mixte paritaire, et le Gouvernement s'en félicite,

Je pense notamment à l'amendement que vous avez accepté de voter prévoyant de débloquer 500 millions d'euros pour financer l'appel à projets pour les industries du futur. Je pense au fonds de participation que nous pouvons encore mobiliser, y compris dans le cadre du plan de relance, 20 milliards d'euros ayant été votés dans le PLFR 2. L'ensemble des dispositions nécessaires au financement du plan de relance devront évidemment être complétées dans le PLF pour 2021 et, si nécessaire, dans le PLFR de fin de gestion.

la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020. J'observe que c'est la deuxième fois

Cette seconde CMP conclusive traduit sans doute l'esprit de responsabilité du Parlement et confirme la capacité de dialogue et d'écoute des deux rapporteurs généraux, Albéric de Montgolfier et Laurent Saint-Martin, que je tiens à saluer pour le travail qu'ils Elle augure aussi- en tout cas nous l'espérons -de belles perspectives pour les séquences budgétaires à venir. Qui sait ? Puisse la volonté de dialogue du Premier ministre se traduire dans les actes ! Nos motifs de satisfaction sont à la mesure des apports du Sénat qui ont été retenus dans le texte final.

L'introduction au Sénat de la clause dite « de retour à meilleure fortune » offrira ainsi une protection précieuse aux départements concernant leurs recettes de DMTO, en leur garantissant qu'ils n'auront à les rembourser que lorsqu'ils auront retrouvé un niveau de droits de mutation équivalent à celui d'avant la crise. C'est une bonne chose. De la même façon, la possibilité offerte de financer des projets couverts par la DETR avec l'enveloppe de 1 milliard d'euros ouverte au titre de la DSIL est une avancée bienvenue. Notre collègue Bernard Delcros en avait émis le souhait en ouverture de la discussion générale. C'est là un beau message adressé à l'échelon départemental, qui, tout au long de la crise sanitaire, a su répondre avec agilité aux besoins exprimés sur le terrain par nos concitoyens. Les membres du groupe Union Centriste se félicitent également de l'inscription dans ce troisième collectif budgétaire des dispositions de la proposition de loi de notre collègue Dominique Vérien, votée à l'unanimité au Sénat, concernant l'élargissement du champ d'application du label de la Fondation du patrimoine. du label de la Fondation du patrimoine. L'extension de ce label aux propriétaires dans des communes allant jusqu'à 20 000 habitants, contre 2 000 habitants jusqu'à présent, permettra de participer à la relance, les bénéficiaires pouvant investir leurs économies d'impôts dans des travaux. L'État en aura forcément un retour grâce à l'impôt sur les sociétés et la TVA qu'il percevra. Concernant Île-de-France Mobilités, l'accord trouvé en CMP n'est certes pas allé jusqu'à renforcer l'acompte versé par l'État. On peut le regretter, mais il est vrai que nous partions de zéro dans le PLFR initial. L'Assemblée nationale a su étendre le bénéfice du prélèvement sur recettes à l'établissement public francilien. La CMP a par ailleurs conservé la modification introduite par le Sénat des paramètres de calcul de la compensation octroyée, laquelle tiendra compte des augmentations de taux intervenues entre 2017 et 2019 pour le financement du passe Navigo. d'Île-de-France Mobilités doit faire l'objet de nouveaux rendez-vous. Le Gouvernement s'y est, je crois, engagé, le rapporteur l'a rappelé il y a quelques instants. Nous serons bien sûr très attentifs au respect de ce point.

Nous serons bien sûr attentifs à la suite qui sera apportée aux demandes de la présidente de la région et d'Île-de-France Mobilités. prospéré à l'issue de la CMP le remboursement anticipé de la TVA acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses d'équipement au titre du FCTVA. Une telle mesure nous semblait vertueuse dans le but évident de relancer l'investissement. Elle aurait immédiatement rendu de la trésorerie aux collectivités et leur aurait donné les moyens d'investir. L'essentiel de nos désaccords a toutefois davantage porté sur des questions de calendrier que sur des sujets de fond. C'est la raison pour laquelle nous sommes confiants alors que se profilent déjà la présentation du projet de loi de finances pour 2021 et la mise en oeuvre du plan de relance.

d'aide à l'embauche des jeunes, qui seront à la rentrée les premiers à pâtir d'un marché du travail devenu malheureusement exsangue sous l'effet de la pandémie. Le compromis trouvé sur ce texte a coïncidé avec l'accord sur le plan de relance européen, dont nous nous félicitons, accord obtenu quelques heures seulement avant la réunion de la CMP. L'expérience du confinement aura peut-être ceci de positif qu'elle accélérera la solidarité et le rapprochement entre les peuples européens. Souhaitons-le en tout cas. La façon dont nous allons relever les défis auxquels nous confronte le covid-19, en particulier d'un point de vue budgétaire, déterminera le devenir de notre pays, comme celui de nos principaux partenaires.

Or, à l'occasion de ce troisième projet de loi de finances rectificative, ni le Gouvernement ni la majorité sénatoriale n'ont fait le choix d'un véritable « budget de combat », protecteur des plus faibles, de nos entreprises, de nos collectivités et de nos territoires. C'est une erreur stratégique majeure d'attendre la rentrée pour lancer un plan de relance et le traduire dans le projet de loi de finances pour l'année 2021. Nous avons pourtant écouté le Président de la République nous dire le 14 juin dernier que près de 500 milliards d'euros auraient été engagés.

Vous trompez les Français sur l'ampleur et la réalité des moyens mis en oeuvre pour lutter contre la crise économique, sociale et écologique. Vous sacrifiez certains secteurs d'activité de notre pays, en arguant faussement de la relance. Mais de quelle relance s'agit-il ? Et avec quels moyens ? de la culture, du tourisme, du BTP et de tant d'autres secteurs qui n'ont toujours pas reçu de réponse politique et budgétaire satisfaisante ? Nous assistons à des stratégies à faire reposer une large partie des conséquences de la crise sur les collectivités territoriales, sur les acteurs économiques et sur les Français eux-mêmes, indistinctement. Nous aurions trouvé équitable que ceux qui ont les moyens de contribuer le fassent à la hauteur de leurs capacités en revenus et en patrimoine. C'est une question financière, mais c'est aussi et surtout une question politique de cohésion sociale. Non ! Tel était le sens des amendements que nous avions déposés tout au long de la procédure parlementaire et qui, malheureusement, pour des raisons idéologiques, n'ont pas été retenus. Même si nous avons, dans un premier temps, obtenu des avancées et une meilleure compensation, pour les collectivités de métropole et de l'outre-mer, des charges liées à la crise, même si nous avions obtenu de quoi sauver les autorités organisatrices de la mobilité, notamment Île-de-France Mobilités, même si nous avions obtenu une taxation plus appropriée des tels qu'Amazon, afin de restaurer une concurrence loyale dans le commerce, après un confinement très déstabilisant, même si nous avions arraché

preuve s'il en est que, en matière d'écologie, les actes du Gouvernement ne suivent pas les mots du Président de la République. Enfin, le choix d'un financement global de ce budget par la dette, sans remise en cause d'une fiscalité avantageuse pour les Français les plus aisés, n'est pas acceptable. Pour ces raisons, nous n'avons pas pu voter ce texte, insuffisamment nous. Mes chers collègues, nous sommes désormais appelés à nous prononcer sur le texte issu de la commission mixte paritaire, qui a largement remis en cause le texte voté par le Sénat, puisque, parmi tous les amendements proposés par notre groupe, un seul, qui tend à conforter le soutien des collectivités locales aux associations impactées par la crise, a été sauvé. Nous ne comprenons pas l'accord qui a été trouvé entre les deux assemblées, dès lors que de nombreux amendements adoptés à une grande majorité, voire à l'unanimité du Sénat dans sa diversité n'ont pas été retenus par la commission. par la commission. Le Sénat n'a pas joué son rôle de défenseur des collectivités et des territoires, comme en atteste le sort réservé aux articles 5 et 6 du texte portant sur les soutiens aux collectivités territoriales et aux territoires ultramarins, fortement affectés par la crise sanitaire. Je m'inquiète d'ailleurs du sort qui sera réservé à Île-de-France Mobilités, à la suite du recul de la majorité sénatoriale. D'une manière plus générale, je m'inquiète de l'incapacité du Gouvernement à comprendre le rôle que peuvent jouer les territoires dans l'accompagnement social des populations qui souffrent et souffriront et le potentiel économique et écologique de ces territoires. Nous considérons que le seul chemin possible passe par la justice fiscale et sociale.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général de la point final d'une session très particulière, ces conclusions de la CMP sur le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 appellent quelques commentaires. Je salue d'abord l'esprit de responsabilité des membres de la commission mixte paritaire, qui, comme lors du deuxième collectif d'avril, ont su trouver un accord sur un texte commun, préservant ainsi certains apports du Sénat, tout en garantissant une adoption consensuelle et diligente, alors que l'urgence de la situation

de 40 milliards d'euros par rapport au PLFR 2 voté en avril. On peut toujours ressentir une certaine frustration à l'issue de ces examens très denses dans des délais très resserrés

Le RDSE s'est montré particulièrement engagé tout au long de l'examen du texte, avec un nombre d'amendements s'inscrivant dans la moyenne haute du Sénat, présentés par de nombreux membres de notre groupe sur des sujets très diversifiés, à l'image de l'attention que nous portons aux nombreux secteurs touchés par la crise actuelle. Je me félicite en particulier de l'adoption par la Haute Assemblée de l'amendement présenté par mon collègue Éric Gold et l'ensemble du groupe visant à mieux informer le Parlement sur l'ampleur et les caractéristiques de la fraude au chômage partiel. Pour ce dispositif, salué à juste titre, mais dont le coût pour l'État s'élève à plus de 30 milliards d'euros, il est impératif de s'assurer de la bonne utilisation des deniers publics, par les salariés aussi bien que par les employeurs, sans préjuger la bonne foi des uns et des autres. Si, hélas, peu de ces modifications sont restées dans le texte de la CMP, on peut tout de même se féliciter, notamment, du maintien de la suppression de l'article 4 , qui aurait eu des conséquences fâcheuses pour le financement des chambres de commerce et d'industrie. Je souhaite également relayer l'inquiétude actuelle quant aux pertes de recettes des collectivités territoriales baisse des DMTO pour les départements, de la TVA et d'autres impôts économiques pour les régions et de différentes recettes fiscales pour les communes et les intercommunalités. Je salue toutefois les mesures fortes prises par le Gouvernement, à hauteur de 4,5 milliards d'euros, pour les soutenir. Il sera difficile à court terme d'évaluer l'impact de ces aides, tant les finances locales sont un domaine complexe et les situations différentes d'une collectivité à une autre. Espérons que ces mesures suffiront Enfin, je ferai une remarque sur l'article 18 de ce projet de loi, relatif aux exonérations. Bien qu'il ait donné lieu à de nombreux amendements et réponde à de réelles difficultés rencontrées par les entreprises, aurait eu davantage sa place dans un budget rectificatif de la sécurité sociale. Si cette discussion est la dernière avant la suspension des travaux pendant l'été, gageons qu'elle ne sera pas, tant la dernière de l'année sur l'évolution de la situation économique et budgétaire. Sans anticiper le débat d'orientation qui suivra, je tiens, au nom d'un groupe engagé en faveur de la construction européenne, à saluer également l'accord historique trouvé à Bruxelles en début de semaine sur un programme de relance économique au niveau de l'Union. Bien évidemment, nous devrons suivre de près les détails de la mise en oeuvre et le processus de ratification. En conclusion, j'indique que le groupe du RDSE votera en faveur de l'adoption de ces conclusions.

le Sénat, en changeant le mode de calcul, c'est-à-dire en prenant l'année 2019 pour référence et non plus la moyenne des trois dernières années, a ajouté 200 millions d'euros aux 450 millions d'euros introduits par Laurent Saint-Martin

de ce projet de loi de finances rectificative. Je citerai les 200 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence, l'aide de 200 euros pour les jeunes de moins de 25 ans qui bénéficient de l'APL (aide personnalisée au logement), soit 400 000 d'entre eux, et l'indemnisation pour les professionnels libéraux qui auraient été contaminés par le covid et qui n'ont pas les assurances

les jalons de la relance : transition écologique, transition numérique, emploi des jeunes, culture et solidarité. Même s'il y a encore du pain sur la planche, je me réjouis que nous ayons pu dépasser un certain nombre de clivages et obtenir, pour la troisième fois, un accord sur un projet de loi de finances rectificative. Notre groupe

La pandémie de covid-19 a rebattu les cartes avec l'irruption du fameux « quoi qu'il en coûte ». Mais c'est un euphémisme que de dire que les résultats de la commission mixte paritaire sont pour le moins décevants. Un constat s'impose néanmoins : au-delà de nos divergences politiques, la crise sanitaire a laissé la place à une crise économique et, désormais, à une crise sociale. Comment trouver les leviers pour relancer notre pays avec une économie quasiment à l'arrêt et un État qui a organisé lui-même son impuissance au gré des privatisations et des libéralisations ? Dans le cadre de ce troisième projet de loi de finances rectificative, majorité sénatoriale et majorité présidentielle ont avancé main dans la main ... Non ! ... pour rejeter toutes les mesures de justice sociale et, surtout, fiscale que nous avions proposées. En accord avec cette politique libérale, il est encore et toujours refusé de toucher à la fiscalité des plus aisés ou de demander des contreparties aux entreprises soutenues par l'État. Vous avez rejeté la taxe sur les Gafam les 150 millions d'euros visant à abonder la recherche scientifique, pourtant indispensable dans le contexte actuel. Vous avez même rejeté une mesure de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, pourtant grande cause nationale de ce quinquennat, en refusant de sanctionner les entreprises ne respectant pas l'égalité salariale par l'interdiction d'exonération de cotisations sociales. La droite refuse de mettre à contribution les 1 % les plus riches qui accumulent des richesses indécentes, tandis que la majorité de nos concitoyens se serre de plus en plus la ceinture. Vous pouvez sourire, mais le débat sur la gratuité des masques n'est pas le fruit du hasard, mes chers collègues. Un groupe de 83 millionnaires a rédigé une lettre, dont je vous cite un extrait : « Les chefs de gouvernement doivent prendre la responsabilité de lever les fonds dont nous avons besoin et les dépenser équitablement pour financer adéquatement nos systèmes de santé, les écoles et la sécurité une augmentation permanente des taxes sur les plus fortunés de la planète, des gens comme nous. Je regrette que l'accord trouvé lors du sommet européen extraordinaire sur la relance de l'Union européenne, que notre Président a tant vanté, n'ait absolument pas repris cette proposition faite par les millionnaires eux-mêmes. Au contraire, on nous explique qu'il faut augmenter la CRDS et la CSG, pour les retraités, les salariés et les assurés sociaux, ou encore raboter les salaires ! Et pourquoi pas travailler plus pour gagner moins ? Lors de la commission mixte paritaire, la droite sénatoriale et le Gouvernement sont tombés d'accord ... Non ! ... - Roger Karoutchi en est un illustre témoin -, s'ils ne l'étaient pas déjà avant. Quand le Sénat adopte des contreparties écologiques et salariales sur les aides aux entreprises, le Gouvernement met son veto. L'argent magique est de retour, mais seulement pour les entreprises, qui conservent leur droit inaliénable à licencier et à polluer.

Le compte n'y est pas ! Nous voulons maintenant des actes, du sonnant et du trébuchant pour aller vers la sobriété énergétique. Pour les collectivités territoriales, les concessions de la majorité présidentielle sont insuffisantes. La clause de sauvegarde pour le bloc communal, mesure phare du plan de soutien aux collectivités, demeure incomplète. La clause de « retour à bonne fortune » concédée aux départements est un moindre mal. Alors qu'il fallait engager 7,5 milliards d'euros pour compenser les pertes et redistribuer à tous les niveaux des collectivités territoriales, on nous propose seulement 4,5 milliards d'euros, soit 3 milliards de moins 3 milliards de moins pour l'investissement et les services publics, qui pourtant bénéficient tant aux citoyens qu'aux entreprises. Il faut d'autres réponses, inédites et ambitieuses, et ambitieuses, permettant de renouer avec la proximité et la présence publique, pour assurer un partage des richesses et une redistribution basée sur la solidarité et l'unité d'une République des biens communs.

Face à la crise, face à une situation que nul ne pouvait envisager il y a seulement six mois de cela, nous avons fait le choix collectif d'activer la solidarité nationale pour sauver notre économie, et ce par-delà les clivages partisans. Les décisions votées au cours des trois PLFR pour 2020 sont lourdes de conséquences. Nous aurons l'occasion d'y revenir en détail tout à l'heure, lors du débat sur l'orientation des finances publiques. Je me contenterai pour l'instant de revenir sur les principales mesures introduites par le PLFR 3. Les collectivités locales se sont enfin trouvées au coeur de nos travaux. Elles n'avaient jusqu'à présent fait l'objet que de mesures éparses et ponctuelles, alors même qu'elles prenaient les devants pour inventer des solutions aux problèmes de leurs administrés. Les réponses que nous leur apportons avec ce texte sont placées sous le signe de l'efficacité et du pragmatisme. Ces mesures permettront ainsi aux collectivités de mieux encaisser la crise économique et même de concourir activement à l'effort de relance. Je pense notamment à la clause de « retour à meilleure fortune » pour les pertes de recettes des départements. Cette disposition, introduite par le Sénat et conservée dans le texte issu de la CMP, était très attendue par les élus locaux. de même pour la possibilité laissée à certaines collectivités de procéder à des dégrèvements de CFE ou à des exonérations temporaires de taxes de séjour en 2020. Il s'agit d'un levier utile mis à leur disposition, dont elles sauront faire usage. Je regrette à cet égard que la commission mixte paritaire n'ait pas retenu le report de la date limite pour voter de tels dégrèvements. Notre groupe avait déposé plusieurs amendements dans ce sens. C'était finalement la date du 15 septembre qui avait emporté l'adhésion de notre assemblée. Avec le retour à la date du 31 juillet, décidé en commission mixte paritaire, nous ne laissons aux collectivités guère plus qu'une petite semaine pour voter des mesures importantes à destination des entreprises et de leurs territoires. Je crois qu'un délai supplémentaire aurait été le bienvenu. Nous risquons, ce faisant, d'envoyer un message négatif aux élus locaux : ce sont les collectivités qui doivent s'adapter aux contraintes de Bercy, et non l'inverse Notre groupe avait également fait adopter un amendement permettant le remboursement des achats de masques réalisés par les collectivités à partir du 1mars. Cette disposition n'a malheureusement pas été retenue dans la version finale du texte. Là encore, nous aurions pu envoyer un message positif aux élus locaux en reconnaissant leur implication dans la crise. Au-delà des collectivités territoriales, ce troisième projet de loi de finances rectificative amplifie les mesures d'urgence pour soutenir notre économie. Elles étaient également très attendues par nos entrepreneurs. Je pense au chômage partiel, aux allégements de charges ou encore au fonds de solidarité pour les entreprises. Le Sénat a également été à l'initiative d'une mobilisation de crédits supplémentaires pour faire face à l'urgence de la situation. Il y va ainsi des moyens alloués à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. En tant que sénatrice d'Île-de-France, j'y suis particulièrement attentive. Je pense également aux investissements industriels, mais aussi et surtout à l'augmentation des crédits consacrés à l'apprentissage.

je tiens à dire un mot d'un secteur qui souffre encore énormément de la crise. Indéniablement, la culture demeure le parent pauvre de la relance qui s'amorce à peine. Je crains que les dispositions finalement retenues ne soient encore très en deçà des attentes. Nous devrons nous en souvenir à l'automne. ce dernier plan de sauvetage précède le plan de relance tant attendu. Au-delà de la question des véhicules législatifs adaptés, nous ne devons plus tarder pour engager vigoureusement la relance. La conclusion de l'accord européen doit nous conforter dans notre détermination. Nous avons obtenu, grâce à la solidarité de nos partenaires européens, les garanties nous permettant de ne pas revoir nos ambitions à la baisse.

à celles de l'Assemblée nationale -, et troisième conclusion positive d'une commission mixte paritaire ! Cela vous montre une nouvelle fois que nous savons être constructifs et pragmatiques quand il s'agit de répondre à l'urgence économique et d'agir dans l'intérêt général.

bien que nous déplorions que le taux de remise ne soit que de 50 % et non pas de 70 %, comme nous l'avions plaidé, pour les plus petites entreprises, celles de moins de 50 salariés. Je pense à la hausse des crédits pour le très haut débit. Je pense également à l'aide au recrutement en contrat d'apprentissage d'étudiants,

Nous acceptons l'accord trouvé en commission mixte paritaire, car il convient de répondre à l'urgence. Mais nous serons très vigilants dans le cadre des textes qui nous seront présentés à l'automne.

pour le transport public quotidien de 5 millions d'usagers en Île-de-France, vous mégotez, pour n'indemniser ni la région, ni la SNCF, ni la RATP.

Monsieur le ministre, vous voulez relancer le

la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

ainsi que les dispositifs permettant de dégager des recettes fiscales et domaniales pour les collectivités territoriales, en métropole comme en outre-mer, avec 2 milliards d'euros d'avance aux collectivités territoriales pour soutenir les départements, dont certains sont particulièrement affectés par des baisses de DMTO. La mission « Relations avec les collectivités territoriales 1 milliard d'euros en autorisations d'engagement au titre de la DSIL et de la DETR, en soutien aux investissements portés par les collectivités territoriales pour aider l'artisanat du bâtiment et l'ensemble du secteur du BTP. Naturellement, le plan d'urgence face à la crise sanitaire atteint

Le scrutin est clos.

la maîtrise de la dépense et de la dette publiques et une application rigoureuse du principe de sincérité budgétaire, qui s'applique autant à nos prévisions qu'à la budgétisation des dépenses. Il ne faut pas négliger le rôle joué par cette bonne gestion dans notre capacité à gérer la crise. Les efforts conduits depuis trois ans ont permis de sécuriser nos marges de manoeuvre pour faire face à des dépenses imprévues et exceptionnelles qui ont été et qui sont encore nécessaires. Les réformes que nous avons menées ont grandement participé à cet état de fait, d'abord par la baisse inédite des prélèvements obligatoires, qui va se poursuivre, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français et de la compétitivité à nos entreprises. J'ai ainsi à l'esprit la suppression de la taxe d'habitation, qui se poursuivra au rythme annoncé,

Ce sont ces réformes qui ont permis de faire passer le taux de prélèvements obligatoires par rapport au PIB de 45,1 % en 2017 à 44,8 % en 2018 et à 43,8 % en 2019, un taux de prélèvements obligatoires que nous voulons préserver. La progression des dépenses a été maîtrisée, notamment grâce à des réformes structurelles dans le champ de la politique du logement, de l'emploi et de l'audiovisuel public. Les administrations locales, qui, nous le savons, font face à des responsabilités croissantes, se sont également engagées dans cet effort commun de maîtrise des finances publiques. Ainsi, les collectivités et les organismes locaux présentent depuis quelques années un solde excédentaire.

puisque le déficit de l'an dernier avait même été réduit à 1,9 milliard d'euros, son niveau le plus faible depuis le début des années 2000. Enfin, la qualité de la gestion publique a été améliorée grâce au travail de sincérisation des prévisions établies en loi de finances initiale. La sincérité s'est accompagnée d'un plus grand respect des autorisations parlementaires, à l'instar des deux derniers budgets rectificatifs. Nous n'avons ainsi pris aucun décret d'avance au cours des deux derniers exercices, une méthode dont nous souhaitons poursuivre en oeuvre. En matière de gestion des finances publiques, des améliorations sont évidemment toujours possibles. La Cour des comptes a récemment souligné, dans son rapport sur l'évolution des finances publiques, la nécessité de mener une nouvelle réflexion sur les modalités de leur pilotage pour l'avenir, dans un contexte bouleversé par la crise sanitaire et par ses conséquences économiques et financières.

La crise sanitaire nous a en effet conduits à agir vite et à prendre des décisions fortes en faisant passer la santé de nos concitoyens au premier rang des priorités. En 2020, ce sont ainsi 8 milliards d'euros de dépenses de santé supplémentaires qui ont été mobilisés supplémentaires qui ont été mobilisés pour financer des commandes massives de médicaments, de respirateurs ou de masques, mais aussi pour le versement de primes, le paiement d'heures supplémentaires ou encore le versement d'indemnités journalières. L'arrêt de l'activité a bouleversé nos entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, ainsi que leurs salariés. Nous les avons aidées, et nous devons redoubler d'efforts pour les accompagner, en particulier, le soutien massif à l'emploi, grâce au financement de l'activité partielle, qui représente aujourd'hui un total de 31 milliards d'euros, et le fonds de solidarité, destiné à venir en aide aux entreprises les plus vulnérables et qui a été étendu dans le PLFR 3 pour représenter plus de 8 milliards d'euros. Par ailleurs, l'État s'est placé en situation d'assureur en dernier ressort de l'économie par la garantie des prêts aux entreprises qui en avaient besoin ; nous avons également mis en place un système de report d'échéances de paiement de prélèvements obligatoires, dont certains feront désormais l'objet d'annulations définies par l'article 18 du PLFR que vous venez d'adopter. Nous avons aussi travaillé à rembourser de manière anticipée les crédits d'impôt et nous avons abondé le compte « Participations financières de l'État » à hauteur de 20 milliards d'euros pour nous permettre de prendre des participations dans des entreprises stratégiques qui auraient besoin de cette intervention pour être pérennisées. Il faut aussi souligner que le confinement a exacerbé les disparités qui existaient au sein de notre société. Il était donc de notre devoir d'assurer, en complément des actions déjà menées, un soutien pour les plus fragiles. C'est la raison pour laquelle nous avons prolongé les revenus de remplacement, différé de quelques mois l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage, mais aussi distribué une prime exceptionnelle aux foyers les plus fragiles et les plus précaires, octroyé une aide supplémentaire pour les jeunes ou pour les étudiants et mis en place des dispositifs d'aide sociale, de chèques services pour l'alimentation ou pour l'hygiène, afin d'apporter une aide nécessaire à ceux qui en avaient le plus besoin. L'ensemble de ces mesures sanitaires, économiques et sociales, ainsi que les garanties apportées par l'État représentent au total 470 milliards d'euros, consacrés à lutter contre la crise et ses conséquences. était de notre devoir d'être à la hauteur des enjeux de cette crise sanitaire, et la dégradation de nos finances publiques était évidemment inéluctable. Personne, à mon sens, n'aurait pu procéder autrement. À ce stade, nos prévisions économiques permettent d'estimer un impact de la crise sur les finances publiques. Ainsi, le solde public pourrait s'établir à moins 11,4 % du PIB en 2020, contre moins 2,2 % dans la loi de finances initiale. Le solde structurel serait en revanche stable, à moins 2,2 %, puisque les effets de la crise revêtent un caractère exceptionnel, que nous devons préserver. La dette, elle aussi, atteindra un niveau record, à 121 % du PIB, mais, malgré cela, nous continuons à jouir de la confiance de nos créanciers, notre crédibilité sur les marchés venant aussi du sérieux de notre gestion. On mesure à quel point cela est essentiel. Nos finances publiques sont utilisées massivement comme instrument de lutte face à la crise. Nous menons une action forte, à la fois ciblée et contracyclique, et nous continuerons à le faire dans les prochains mois. Pour les deux ans à venir, la priorité sera la relance.

Ces prévisions sont encourageantes, mais elles restent très incertaines. La reprise de l'activité demeure dépendante de la situation sanitaire, et la crise a aussi pu entraîner des changements structurels dans les entreprises, dont nous ne mesurons sans doute pas encore toutes les conséquences.

Afin de conforter la croissance, nous devons porter un plan de relance pour notre tissu économique, dont les mesures seront au coeur du projet de loi de finances pour 2021, qui sera présenté dans les prochaines semaines. Elles trouveront leur place dans une mission spéciale de relance

sera accompagné- c'est une première -d'une budgétisation verte, qui nous permettra de mesurer l'impact environnemental de notre action. Cette innovation méthodologique offrira une offrira une réelle visibilité des effets de l'action publique en matière d'environnement. C'est la première fois qu'un pays se prête à cet exercice à l'échelle de son budget national. Les mesures dédiées à la relance seront donc regroupées dans une nouvelle mission du budget de l'État, qui sera temporaire et se trouvera en dehors du périmètre de la norme de dépenses pilotables, pour faciliter la lecture de notre action. Chaque politique publique portera ainsi les crédits du budget général et du plan de relance. Le budget pour 2021, hors plan de relance, dont les premiers équilibres vous sont présentés dans le document qu'il est convenu d'appeler le « tiré à part », confirme notre sérieux et notre engagement budgétaire. Avec une progression des dépenses pilotables de l'État de 2,6 %, soit 7,2 milliards d'euros, le Gouvernement a choisi de construire un budget qui reprend la trajectoire triennale comme point de référence, actualisée des priorités nouvelles nées de la crise et des engagements pris par le Gouvernement et le Président de la République. Ainsi, à titre d'illustration, les armées, qui ont bénéficié d'un renforcement sans précédent de leurs moyens depuis 2017 avec une augmentation de 5,2 milliards d'euros en trois ans, verront leur budget doté de 1,7 milliard d'euros supplémentaires en 2021, notamment en faveur de la défense spatiale. Les moyens de la justice seront augmentés, grâce à une progression de son budget de 6 %. Notre ambition est aussi de continuer à investir dans les savoirs et les compétences. Notre action doit notamment permettre aux jeunes de construire leur avenir sereinement et de bénéficier d'opportunités professionnelles, tout en participant à la construction de l'avenir de notre pays. C'est la raison pour laquelle le budget de l'éducation nationale progressera de 1,3 milliard d'euros et le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche de plus de 300 millions d'euros. Toujours pour financer nos priorités, les crédits alloués à la transition écologique s'élèveront à plus de 26 milliards d'euros, soit une hausse de 550 millions d'euros, auxquels s'ajoutera une enveloppe majeure du plan de relance, puisque nous avons la volonté que celui-ci soit le plus vert possible.

le budget dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes augmentera de près de 40 % pour répondre aux priorités et aux engagements pris. Ces orientations doivent servir de cadre à la discussion qui commence aujourd'hui. Je sais votre engagement en faveur de l'intérêt général et des comptes publics et je connais, d'expérience, la qualité de nos échanges. Je suis convaincu qu'ils nous permettront de construire ensemble un budget susceptible de nous remettre sur le chemin de la croissance et de l'emploi. J'insiste sur le fait que ce budget général sera

de manière que, lorsque nous aurons atteint le niveau de production de richesses qui était le nôtre avant la crise, nous retrouvions des conditions de poids des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques qui ne soient pas dégradées par rapport à la période précédant la crise, mais que nous continuions, au contraire, à bénéficier des efforts faits, en allant plus avant en la matière. La parole est

Je souhaite néanmoins appeler votre attention sur un point de vigilance qui concerne l'effet de la crise sur le PIB potentiel. En effet, le Gouvernement continue de faire l'hypothèse que la crise n'aura aucun effet sur le PIB potentiel et que la perte d'activité sera intégralement rattrapée. Or il s'agit malheureusement d'une hypothèse optimiste, compte tenu de l'ampleur des défaillances d'entreprises et de la hausse du chômage anticipées, d'une part, et de l'expérience des récessions précédentes, d'autre part. La plupart des organisations internationales et des instituts de conjoncture ont ainsi retenu une hypothèse plus prudente que le Gouvernement. d'illustration, la Banque de France table sur une perte définitive de PIB potentiel de l'ordre de 1,5 point, mais considère que la croissance potentielle ne serait en revanche pas affectée, tandis que la Commission européenne a d'ores et déjà revu à la baisse sa prévision de croissance potentielle. Il serait souhaitable à l'avenir de retenir un scénario plus prudent, selon lequel la crise aurait un effet sur le PIB potentiel, sans nécessairement grever la croissance potentielle. Cela permettrait, notamment, de porter une appréciation plus prudente sur la situation structurelle des comptes publics. Sur le plan budgétaire, le Gouvernement anticipe un recul du déficit public à 5,5 % du PIB en 2021, après le chiffre

Le ratio d'endettement diminuerait légèrement pour atteindre 117,5 % du PIB, après 120,9 % en 2020, du fait de l'effet dénominateur lié au rebond de l'activité. Si le Gouvernement ne nous donne pas d'indication sur le niveau du déficit structurel, il s'agit, là encore, d'un point de vigilance. Comme je l'ai rappelé maintes fois dans le cadre du débat sur le PLFR 3, les mesures de soutien et de relance de l'économie doivent être immédiates,

Si le rapport préalable au DOFP intervient sans doute un peu trop tôt pour que le Gouvernement puisse clarifier ses intentions en la matière, il est impératif que le projet de loi de finances pour 2021 comporte un volet pluriannuel permettant de donner de la visibilité à la stratégie de moyen terme du Gouvernement en matière de finances publiques.

Premièrement, la poursuite du soutien au tissu productif en 2021, dès lors que celui-ci ne devrait pas se traduire par une hausse de la charge de la dette à court terme et permettrait de préserver le potentiel de l'économie française. Il serait contre-productif de chercher à augmenter les impôts ou à diminuer certaines dépenses tant que le rattrapage du terrain perdu pendant le confinement n'est pas achevé. Deuxièmement, un effort continu de redressement des comptes publics à moyen terme, fondé sur la maîtrise de la dépense publique, afin de retrouver des marges de manoeuvre en vue des futures crises et de nous prémunir contre le risque de remontée des taux d'intérêt.

Les principaux chiffres sont impressionnants : une forte augmentation des dépenses d'assurance maladie, de l'ordre de 8 milliards d'euros, qui pourrait faire progresser l'Ondam d'environ 6,5 % en 2020 ; une très forte contraction des recettes, à la fois de l'érosion de l'assiette des cotisations et des contributions sociales et des dispositifs de reports massifs utilisés par les employeurs pendant le confinement ; une dernière prévision officielle de déficit consolidé

touchée par le traditionnel effet de ciseaux sur ses recettes et ses dépenses en cas de crise économique. Ainsi, alors que cet organisme devait renouer avec l'équilibre cette année,

jusqu'à 63 milliards d'euros à la fin de l'année, ce qui poserait un problème majeur pour son apurement. Dans un débat sur l'orientation des finances publiques, il me semble que nous devons tirer quelques enseignements de cette situation. Tout d'abord, constatons ensemble que, toutes proportions gardées, ce n'est pas la trajectoire financière de 2020 qui pose problème, mais surtout l'insuffisant rétablissement des comptes sociaux avant la crise.

En revanche, au vu de la nature des dépenses de protection sociale, il revient à chaque génération de s'autofinancer en la matière, sans reporter le poids de ses dépenses sur les générations suivantes- on ne cesse de le répéter, mais ce n'est pas aujourd'hui totalement acté ... De fait, l'histoire des finances sociales montre une très grande difficulté des pouvoirs publics, quelle que soit la législature, à parvenir à cet équilibre des comptes, qui implique

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous devrons avoir le courage de rompre avec cette logique, une fois sortis de la situation économique actuelle. Nous devons assumer la nécessité d'équilibrer nos comptes sociaux, au risque de rompre la confiance, déjà fragilisée, de nos concitoyens dans la pérennité de notre système social. C'est la raison pour laquelle le Sénat a proposé, dès l'examen du projet de loi organique relatif à la dette sociale et à l'autonomie, l'instauration d'une règle d'or.

de base et du FSV par périodes de cinq ans, voire dix ans en cas de circonstances exceptionnelles. Je ne vous cache pas, monsieur le ministre, que nous avons été surpris de l'opposition du Gouvernement à l'instauration d'un tel cadre, alors même que notre

part, s'accordait avec la volonté exprimée ici même par le Premier ministre le 16 juillet dernier : faisant observer que, « consolider notre modèle de protection sociale, c'est aussi prendre les mesures nécessaires pour assurer sa pérennité », il a jugé nécessaire », il a jugé nécessaire de demander aux partenaires sociaux de « se saisir, avec l'État, des questions liées à l'équilibre de l'ensemble des régimes de protection sociale ». Si je comprends bien, cela correspond tout à fait à notre proposition de règle d'or Face à ces orientations pour le moins contradictoires, peut-être pourriez-vous, monsieur le ministre, nous préciser la trajectoire financière qu'envisage le Gouvernement pour la sécurité sociale pendant et après la crise actuelle.

tient à notre surprise et à notre forte désapprobation face au refus réitéré du Gouvernement de déposer un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, alors que pas moins de trois collectifs budgétaires ont été débattus- le dernier, ici

dans la mission « Solidarité, intégration et égalité des chances » et appelons de nos voeux la rebudgétisation, au sein de cette même mission, du financement des différentes agences sanitaires financées par la sécurité sociale, à commencer par l'Agence nationale de santé publique.

Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, le débat que nous tenons aujourd'hui, en application de l'article 48 de la LOLF, a pour objet de préparer l'examen du projet de loi de finances ; il s'appuie sur les informations délivrées par le Gouvernement à cet effet. Il ne porte toutefois pas sur le seul budget de l'État,

des finances publiques est le seul moment, très elliptique, d'un débat consolidé sur nos finances publiques, alors que l'on voit très clairement, en prenant les seuls exemples du chômage partiel, des exonérations de charges ou du Ségur de la santé, que les problématiques sont partagées. Il en va de même pour les relations financières de l'État avec les collectivités territoriales. Cette année est particulière, en ce qu'elle marque plutôt une désorientation qu'une orientation de nos finances publiques- pardonnez-moi ce mot d'esprit ... Le Gouvernement, en septembre dernier, donc par temps calme, avait préféré reporter l'actualisation de la loi de programmation 2018-2022, pourtant déjà largement obsolète, au motif des incertitudes liées au contexte macroéconomique et à la réforme des retraites. voilà désormais rattrapé par des incertitudes plus grandes encore, qui rendent fragile, sinon illusoire, tout exercice de programmation. De fait, à l'instar du programme de stabilité

Nous avons déjà largement mentionné ces chiffres, ainsi que les mesures prises pour remédier à la crise économique et financière, dans nos débats sur le PLFR 3. J'insisterai donc davantage sur les éléments de débat spécifiques à la préparation

en prendre la mesure pour changer ce qui doit l'être. Tout d'abord, le Gouvernement nous annonce « un rebond économique fort en 2021 », soit une croissance de 8 %, « hors effet du plan de relance à venir

prudent. Bref, les prévisions ne valent que pour ceux qui les présentent ... Je pense en particulier aux risques sanitaires, toujours présents, et aux tensions commerciales et internationales. Par ailleurs, malgré ce rebond, le PIB demeurerait en 2021 inférieur d'environ 4 % à son niveau de 2019. Le Gouvernement compte s'appuyer en 2021 sur le plan de relance européen pour financer une grande partie des mesures qu'il présentera cet automne. L'accord trouvé en début de semaine au Conseil européen doit, bien sûr, être salué, même s'il est moins ambitieux qu'envisagé, puisque les subventions sont ramenées de 500 milliards à 390 milliards d'euros.

La France obtiendrait 40 milliards d'euros, dont une part importante serait versée en 2021 et 2022. Il importera que les procédures d'évaluation par la Commission européenne et d'approbation par les États membres soient suffisamment souples et efficaces pour que ces moyens supplémentaires,

au sujet d'une relance verte. Au-delà de la communication prévue, nous serons vigilants sur la réalité des moyens mobilisés pour la transformation de notre économie, mais aussi pour le soutien aux ménages, qui seront durement touchés par la crise et les licenciements. Enfin, je ne puis pas conclure sans souligner le changement de cap à 180 degrés du Gouvernement en matière d'effectifs publics. qu'une baisse de 50 000 emplois au sein de l'État et de ses opérateurs était annoncée dans la loi de programmation des finances publiques, sur la période 2018-2019 le résultat s'établit plus modestement à 7 148 équivalents temps plein de moins ; et, désormais, le Gouvernement annonce, sans en donner le nombre, des créations d'emploi en 2021, affectées, sauf exceptions justifiées, dans les services départementaux de l'État. Ce matin, Bruno Le Maire a évoqué une « maîtrise de l'évolution de l'emploi public », avec des augmentations d'emplois dans la police, la justice et la santé, mais aussi des réductions d'effectifs dans les secteurs où cela est possible- il a cité le ministère des finances. La crise sanitaire et économique que nous vivons aura le mérite de faire découvrir au Gouvernement l'importance de nos services publics de proximité de la solidarité nationale ... Encore faudra-t-il, plutôt que d'annoncer de nouvelles baisses d'impôts, s'interroger sur les moyens de financer ces services publics, notamment en faisant contribuer ceux qui en ont les moyens. Nous en reparlerons à l'automne

tous aussi aléatoires, dépassés ou provisoires ; je m'en tiendrai à un propos plus général. Le débat sur l'orientation des finances publiques pour 2021 aurait dû avoir pour cadre de référence la loi de programmation des finances publiques pour la période 2018-2022. Celle-ci reposait sur des bases réalistes et intégrait des hypothèses raisonnables sur des facteurs variables. À l'époque de son adoption, à la fin de 2017, nous avions bien noté que, face à des événements conjoncturels imprévus, la trajectoire retenue laisserait peu de marges de manoeuvre pour des initiatives de relance. Personne alors n'avait anticipé le coût budgétaire du mouvement des « gilets jaunes », encore moins celui de la crise sanitaire majeure que nous connaissons ... Face à un choc économique massif, qui aurait sans doute pu être atténué si nous avions maintenu un taux d'activité plus élevé en mars et avril, la réponse du Gouvernement et du Parlement en termes de soutien à l'économie a été à la hauteur des enjeux pour préserver notre appareil productif et nos structures économiques. Au prix, bien entendu, d'un effort budgétaire sans précédent, de 136 milliards d'euros- sans compter les mesures prises au titre du prêt la récession prévue pour 2020, de 11 % du PIB, est supérieure à celles prévues pour l'Allemagne, les Pays-Bas et même, de manière plus surprenante, l'Italie.

-et des entreprises dont le surcroît d'endettement limitera nécessairement les capacités d'investissement. J'insiste sur ce dernier point, car il me paraît sous-estimé par un certain nombre de spécialistes et par le Gouvernement : intégrer dans la structure financière des entreprises

assez complet a été déployé. Sur ces derniers points, le plan de relance de l'automne aura un rôle majeur à jouer pour la capacité de notre économie à rebondir. Face à ces grandes incertitudes, l'objectif raisonnable serait de stabiliser la situation en cantonnant le surplus d'endettement dû au covid-19, amortissable et finançable avec une sorte de « CRDS XXL

pour les élus locaux que nous sommes, ce qui a été perçu comme une innovation pour l'État et a été rendu obligatoire par la LOLF était un rendez-vous bien connu depuis la loi du 6 février 1992. Ce débat d'orientation est, je crois, davantage une consultation du Parlement par le Gouvernement, même si ce dernier a le monopole de la préparation du projet de loi de finances. Je parle de consultation, parce que le Sénat est en prise avec la réalité des territoires, les préoccupations des Français,

Ce débat est l'occasion d'un bilan d'étape des mesures prises par le Gouvernement en ce qui concerne les grandes priorités du quinquennat : 1,7 milliard d'euros par an pour les armées, hausse des crédits des missions « Sécurité » et « Justice » et augmentation des crédits alloués à la transition écologique et aux transports,

prévoyait déjà une avancée majeure, avec l'obligation de ce débat d'orientation budgétaire et les obligations de transparence faites au Gouvernement pour faciliter le contrôle du Parlement, le contexte social et politique de notre pays a changé. Cette année revêt un caractère particulier et montre la difficulté d'articuler programmation pluriannuelle, autorisation annuelle, et gestion infra-annuelle. En trois lois de finances rectificatives, la croissance est passée de 1,3 1,3 % à-11 % du PIB pour 2020, le déficit de 2,2 % à 11,5 % du PIB ... Circonstances exceptionnelles, pourra-t-on dire. Mais, nos débats l'ont montré, ces textes s'inscrivent dans une stratégie de plus long terme, y compris en ce qui concerne les marges de manoeuvre

Quitte à nager à contre-courant, je pense qu'elle est nécessaire et devrait être contraignante pour l'État comme pour le Parlement. Je vois deux options : soit cette programmation s'inscrit dans un mandat politique, en début du quinquennat ; soit elle permet au contraire de sortir du cadre politique en s'inscrivant dans le temps long. La première option nous permettrait de répondre au sentiment chez les Français d'impuissance du politique, qui se réveille notamment en ce moment, où les Français ont l'impression que, lorsque l'État veut, l'État peut, et les arguments budgétaires n'existent plus. La seconde aurait l'avantage de sortir de la logique partisane de la V République, contestée par les Français, et permettrait de travailler à des consensus complexes, mais utiles pour le pays sur le long terme. Elle demanderait aux élus un plus gros effort, tant, nous le voyons sur ces travées, le passé et les quinquennats précédents sont fantasmés, loin de la réalité des chiffres et du vécu social de l'instant. Le débat d'orientation des finances publiques doit aussi être le moment pour le Parlement de donner son opinion sur les choix à opérer pour le prochain budget.

46 milliards d'euros ... Nous avons un modèle à inventer au niveau européen et nous devons investir massivement dans les interconnexions transfrontalières. La souveraineté est aussi numérique : nous avons besoin de systèmes d'exploitation européens.

24 % en 1980 à 14 % en 2007 et à environ 10 % aujourd'hui ; plusieurs millions d'emplois ont été perdus. Il est important que l'État soit au chevet de l'industrie pour éviter la fuite des compétences des territoires. Si l'intervention publique directe peut être justifiée, notamment pour venir en aide à certains secteurs en difficulté, je crois que, là aussi, nous devons rester humbles, compte tenu des échecs passés, sur la capacité de l'État à prévoir les secteurs d'avenir : rappelons-nous le plan Calcul et l'échec de Bull paraît plus que jamais nécessaire : accroître les financements de l'enseignement supérieur et de la recherche, améliorer les liens entre recherche publique et recherche privée, cette dernière étant faible en France alors que notre pays se distingue en matière de recherche fondamentale, rendre la fiscalité plus incitative à la prise de risque, accroître la concurrence en renforçant l'intégration des marchés des biens et services et en réduisant les barrières à l'entrée sur les marchés réglementés. Plus généralement, nous connaissons aussi les déterminants de la croissance : nous devons augmenter le taux d'emploi dans notre pays, notamment celui des seniors, ce qui aura un effet mécanique sur notre PIB potentiel. Monsieur le ministre, chers collègues, sur les grands chantiers de la relance, nous faisons la proposition suivante : que chaque investissement fasse l'objet d'une étude de rentabilité socio-économique, menée par un organisme indépendant du Gouvernement. Notre pays devra investir massivement, mais surtout dans des projets qui auront un effet important sur le PIB potentiel de notre pays. Rendez-vous à la fin de l'été pour le plan de relance

le Président de la République le 12 mars dernier pour évoquer la lutte de la France contre l'épidémie et la crise économique qui en est résultée. Le même jour, Emmanuel Macron a tenu des mots forts, sur lesquels, étonnamment, nous pouvions nous accorder : « Il nous faudra, demain, tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, notre État-providence ne sont pas des charges, mais des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché.

Depuis le mois de mars, nous avons multiplié les dispositifs de soutien d'urgence et de défiscalisation. La situation, à bien des égards, l'exigeait ; c'est pourquoi notre groupe, en responsabilité, a voté ces exonérations de cotisations. que, comme l'a expliqué un de nos collègues samedi soir en s'opposant fermement à la multiplication des ouvertures de crédits, « l'argent gratuit est une illusion ». Dès lors, comment comprendre que le Gouvernement et les majorités parlementaires s'opposent depuis trois mois à ce que l'argent versé aux entreprises s'accompagne d'engagements sociaux et écologiques de ces dernières ? L'exemple de Sanofi est symptomatique du déséquilibre progressif entre capital et travail. L'entreprise pharmaceutique qui, en période de pandémie, a évidemment va supprimer un millier d'emplois en France, tout en continuant à toucher plusieurs centaines de millions d'euros au titre du crédit d'impôt recherche et en ayant versé- au passage -4 milliards d'euros de dividendes, qui sont sortis de l'économie réelle il y a quelques semaines.

L'autre point saillant de l'intervention du 12 mars concerne la prise de conscience de l'urgence d'un réinvestissement massif dans les services publics et les dispositifs de sécurité. Mais, une nouvelle fois, les promesses n'engagent que celles et ceux qui y croient.

Dans un autre domaine, la montagne du Ségur a accouché d'une souris avec une augmentation du revenu des soignants, qui maintient les personnels français sous la moyenne de l'OCDE et qui précarise encore davantage les conditions d'exercice En matière d'éducation, la réussite exceptionnelle au baccalauréat cette année mettra les universités en difficulté : elles seront dans l'incapacité d'accueillir tout le monde. Concernant la sécurité sociale, les mesures les mesures d'urgence prises pour les entreprises ont bien sûr aggravé le déficit. De plus, la création d'une nouvelle branche devrait coûter la bagatelle de 136 milliards d'euros à la Cades. Ce faisant, vous avez d'ailleurs opéré un véritable tour de passe-passe. Vous transférez aux hôpitaux la dette que vous étiez censé leur reprendre ... Faut-il en outre rappeler que la moitié de la dette sociale, que vous ne cessez de dénoncer, est la suite logique, la conséquence mécanique des 66 milliards d'euros d'allégements que vous avez accordés aux entreprises l'an dernier Je pense notamment au remplacement du CICE par la suppression des cotisations à la branche famille, les transformant en une cotisation quasiment symbolique. alimentée par les choix gouvernementaux, sert de justification à toutes les régressions sociales. Je pense par exemple à la réforme de l'assurance chômage ou à celle des retraites, qui revient sur le tapis. C'est cette même réforme qui indexe les pensions sur le niveau du PIB, alors même qu'on voit bien qu'une récession sévère pointe à l'horizon Tout l'édifice de la puissance publique de l'État et des collectivités territoriales est de plus en plus contraint. Monsieur le ministre, reviendrez-vous sur la CAP 2022 ? Conduirez-vous une réforme ambitieuse permettant de reprendre la main sur des pans essentiels à la vie de nos concitoyens ? Où est la mobilisation exceptionnelle promise par le Président de la République ? Bien entendu, lorsque l'on parle d'investissements publics, on nous renvoie à la dette. Mais c'est oublier rapidement que la dette se nourrit autant, si ce n'est plus, des investissements que du manque à gagner fiscal. C'est là un énorme chantier qui doit être mené, car la vérité est bien loin des caricatures qui sont faites d'une France mise à genou à cause de l'impôt. La France se situe derrière le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, la Belgique, la Finlande, la Suède ou encore le Danemark en matière d'imposition sur le revenu. En matière d'imposition sur le travail, elle est quatrième derrière la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. En matière d'imposition sur les sociétés, enfin, elle se situe même sous la moyenne de l'OCDE. Reste enfin la fiscalité des plus hauts revenus, qui ont vu leur taux d'imposition passer de 60 % à moins de 45 % en une cinquantaine d'années. Il existe en la matière des perspectives. Je terminerai en évoquant la réponse européenne. En début de semaine, le plan finalement annoncé se veut bien moins ambitieux que prévu. Surtout, il s'appuie sur les mêmes recettes que celles qui ont affaibli les États : recours accru à l'endettement et engagements structurels le MES. Cette solution ne peut qu'aggraver la crise, priver les États de leurs capacités d'investissement et réduire la voilure des services publics sur le modèle des pays dits « frugaux »- mot à la mode ces temps-ci -, qui ont principalement constitué leur assise financière en devenant des paradis fiscaux au sein de l'Europe- je pense aux Pays-Bas -et en menant un dumping fiscal bien éloigné d'une construction européenne solidaire et rassembleuse. Très bien

Monsieur le président, monsieur le ministre,

Le temps nous est compté pour pousser à fond la transition écologique, mais il nous est aussi compté pour engager notre pays sur la voie du désendettement. Tel est le double défi qui nous attend. Je dis double, car il serait bien irresponsable de vouloir traiter l'un puis l'autre de ces deux aspects sans prospérité économique, pas de transition écologique ambitieuse ; sans priorité écologique, pas de résilience économique et financière. Je le dis au nom de mon groupe : dette publique, dette écologique, même combat ! Il n'y a pas d'alternative. Tel est l'esprit dans lequel nous abordons ce débat d'orientation des finances publiques. la stratégie pour les années à venir, afin de répondre à cet impératif majeur : réduire cette double dette que nous avons laissé enfler durant tant d'années à cause de notre insouciance.

Pareilles mesures s'imposent à nous, dès lors qu'elles ne contredisent pas l'impératif écologique. Nous aurons besoin de toutes nos entreprises pour entamer la relance, de même que pour accélérer la transition écologique. Il s'agit de préserver autant que possible notre tissu économique en attendant les jours meilleurs. La décision prise par le Gouvernement de ne pas augmenter les impôts va dans le bon sens. Nous aurons besoin de capitaux pour innover et inventer les modèles économiques de demain. Nous devons donc continuer à encourager les investissements, que ce soit dans le domaine public ou dans le secteur privé. Mais cet arbitrage fiscal, pour rationnel et stratégique qu'il paraisse, nous oblige. Il nous oblige à réduire de manière draconienne la dépense publique, aujourd'hui supérieure à 60 % de notre PIB et largement au-dessus de la moyenne de la zone euro, sans quoi le rétablissement de l'équilibre budgétaire et la réduction de notre dette publique, sont inenvisageables à moyen terme. Voilà donc le véritable défi sur le plan budgétaire pour les années qui viennent. Bien sûr, nous ne relèverons pas un tel défi en nous contentant d'une approche comptable. Il faudra investir dans une relance qui combine intelligemment écologie et économie, en misant sur une croissance verte. Mais une dette publique au-delà de 120 % de notre PIB n'est pas seulement une réalité comptable. C'est d'abord une réalité qui pèse sur notre souveraineté nationale et compromet notre liberté collective. C'est un fardeau que nous laissons à nos enfants et à nos petits-enfants, alors que nous leur laissons déjà une dette écologique. Il nous appartiendra donc, dans les prochaines années, de leur montrer que nous n'avons pas renoncé à corriger le tir. C'est pourquoi, monsieur le ministre, notre groupe souhaite connaître les grandes orientations que le Gouvernement compte donner à la politique économique, afin de maîtriser la dette publique. Certes, la relance ne fait que commencer, mais il n'est pas envisageable de laisser l'argent public couler à flots, en espérant que la croissance ainsi relancée ne finisse par renflouer les caisses. Il faut prévoir une trajectoire des finances publiques qui soit à la fois raisonnable en termes de discipline budgétaire et ambitieuse en termes de relance économique. Tel doit être l'objectif du Gouvernement, et le Parlement devra le soutenir dans cette démarche de responsabilité. Il s'agit de ramener au plus vite notre pays sur un chemin qui l'expose moins à la volatilité des marchés financiers. Voilà le défi qui nous attend, mes chers collègues. Vous n'êtes pas sans savoir que le débat qui nous occupe aujourd'hui devait initialement se tenir il y a une semaine. Si je fais abstraction des considérations pratiques, je me réjouis que l'ordre du jour ait été ainsi chamboulé. Et pour cause, un événement majeur est survenu dans l'intervalle qui change radicalement les termes de notre débat. Je pense évidemment à l'accord obtenu par le Conseil européen après des négociations marathon. L'étape qui a été collectivement franchie par les Vingt-Sept constitue un moment historique. Nous savons tous le rôle déterminant que la France a joué dans l'obtention de cet accord- le crédit en revient assez largement au Président de la République. La donne a donc changé. Notre pays, qui devrait obtenir près de 40 milliards d'euros de cet accord, a de quoi s'en satisfaire. Cela lui conférera des marges de manoeuvre budgétaires adaptées à la gravité de la situation. Mais c'est surtout le projet européen qui y trouvera un nouveau souffle. Cet accord est le gage d'une intégration renforcée entre nos pays, déjà liés par des relations intenses et étroites. C'est un immense pari que nous faisons ensemble. Je suis persuadée que l'économie de l'Union, malgré toutes ses disparités, repartira de plus belle. Je me permets toutefois d'apporter une touche de réalisme à ce tableau. Je crois qu'il serait dangereux de considérer que l'endettement, parce qu'il a changé d'échelle, a aussi changé de nature. La dette contractée par l'Union européenne devra être remboursée- chacun le sait. Le plan de relance européen est une immense opportunité pour la France, mais, comme toute opportunité, il comporte des risques. Le succès du plan de relance ne tiendra qu'à la possibilité d'une croissance retrouvée dans notre pays et chez nos partenaires. Plus que jamais, les destins de nos nations sont liés par un engagement commun.

Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues,

en 2019, les comptes étaient encore proches de l'équilibre, mais se dégradaient un tout petit peu par rapport à 2018. C'est ce que relève la Cour des comptes. Prenons

l'arme au pied, mais il ne voit toujours rien venir, ce qui est tout à fait insupportable. Alors, vous avez trouvé la solution : c'est le paquet Cades, qui est l'inverse du paquet cadeau, c'est-à-dire que vous emballez le tout sauf que, à la fin, il faut payer ce qu'il y a dedans. Et c'est bien ça le problème

que, un jour, il y ait une vraie crise financière pour engager toutes les réformes. C'est, hélas, souvent ainsi dans ce pays, qui a renoncé. Pour retrouver une trajectoire soutenable,

vous l'avez montré dans votre document, nous sommes totalement à côté de la plaque en 2020 par rapport à la trajectoire initiale. Ce n'est pas supportable. Cette loi de programmation des finances publiques ne fonctionne pas. Il nous faut une

dorénavant une vraie règle d'or pour le budget de l'État : nous n'investissons plus dans ce pays et sommes dopés par des taux d'intérêt bas, qui nous aident en définitive à compenser la hausse de nos dépenses publiques : 2,5 % cette année selon les documents que vous nous avez transmis ce matin. Oui, investir est l'autre

dans un contexte grave, mouvant, exceptionnel, ce qui donne à ce débat une signification toute particulière. La pandémie de covid-19 et le confinement sanitaire engendrent en effet une crise économique d'importance, une récession sévère dans le monde et en France, qui équivaut pour notre pays

Nous courons toujours après la croissance et la pleurons même quand elle est en recul, mais, en 2015, vivait-on réellement moins bien ? Plus grave, le taux de chômage risque de dépasser les 11 % avec une augmentation de la précarité partout en France. Il faudra apporter des réponses rapides pour soutenir nos concitoyens les plus en difficulté. ce sont des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires qui vont être confrontés à la réforme de l'assurance chômage, qui a certes été repoussée pour l'instant, mais qui entrera en vigueur en 2021. Il faut rappeler que la baisse des indemnisations devait concerner au moins 650 000 demandeurs d'emploi et que le durcissement des conditions d'ouverture des droits devait entraîner la radiation de plus de 1,3 million de chômeurs. De surcroît, de nombreuses entreprises, qui, hier, semblaient assurées d'un avenir, baissent aujourd'hui le rideau avec, à la clé, de plus en plus de licenciements. Demain, sans doute, des reprises de dettes, des recapitalisations, des nationalisations seront nécessaires pour sauver les entreprises en difficulté à cause de la hausse prévisible de leur endettement. Pour limiter la casse, le rapport préparatoire au débat sur l'orientation des finances publiques présenté par le Gouvernement fait état d'un budget de relance, dont on apprend qu'il sera dévoilé le 24 août prochain. C'est beaucoup trop tard ! Ce plan contiendrait plusieurs orientations. Il est question de soutenir la reprise de l'activité. Mais de quelles activités parle-t-on ? Des activités polluantes ? Des activités qui soutiennent l'obsolescence programmée ? Aussi, je m'étonne de la distribution massive d'argent public à à certaines entreprises qui produisent seulement 17 % de leurs voitures en France ou d'autres, comme Air France, qui prévoit de supprimer plus de 7 500 postes. Il est aussi question d'accompagner les plus fragiles. Nous avons écouté le Premier ministre et le ministre de l'économie annoncer un plan massif de soutien pour la jeunesse. Soyons plus nuancés : vous avez fait des annonces pour les entreprises, afin de les inciter à recruter des jeunes ; en revanche, aucun filet de solidarité n'est mis en oeuvre pour la jeunesse, qui ne peut bénéficier ni du RSA ni du chômage. À part les repas à 1 euro pour les Crous, il n'y a aucune aide. Tout comme il n'y a aucune ligne budgétaire pour illustrer d'autres dispositifs annoncés. Dans ces conditions, comment y donner du crédit, surtout après la succession de mesures pénalisantes que vous avez mises en place depuis le début du quinquennat ?

de mettre en oeuvre la contemporanéité des aides, heureusement repoussée, qui devait se traduire par une baisse de 1,3 milliard d'euros des APL en année pleine. l'effet cumulé des mesures fiscales et sociales prises en 2018, 2019 et 2020 sur le revenu disponible en 2020 se résume en peu de mots : beaucoup pour les très riches et bien peu pour les plus pauvres. Les gains sont modestes pour environ la moitié des ménages. En revanche, tous les gains se concentrent sur les 1 % des ménages les plus riches, allant même jusqu'à 23 000 euros pour les 0,1 % des plus riches, selon le rapport de l'Institut des politiques publiques. Il est question de renforcer notre souveraineté. Va-t-on racheter la branche stratégique d'Alstom vendue à General Electric, par exemple ? L'État va-t-il prendre sa part dans la reprise de France Rail, ce producteur de rails, qui est le principal fournisseur de la SNCF ? il est question de favoriser la poursuite des transformations structurelles de l'action publique. Jusqu'où va-t-on aller dans le détricotage des services publics ? Nous avons pourtant vu combien nos services publics, notamment l'hôpital public, jouent un rôle essentiel dans notre pays. À y regarder de plus près, vos orientations budgétaires n'offrent pas de grandes surprises. On se contente de colmater les brèches avec des reports de dépenses fiscales et sociales accordées aux entreprises, des facilités ou des garanties d'emprunt qui leur sont proposées. Est-ce suffisant ? Je ne le pense pas. Pourtant, certains de nos partenaires européens se sont engagés dans des dynamiques nouvelles : l'Espagne vient de mettre en oeuvre un revenu de base en moins d'un mois ; l'Allemagne a présenté son plan d'urgence le 3 juin

Depuis plusieurs mois, le gouverneur de la Banque de France sonne l'alarme, jugeant la croissance de la dette privée trop forte et en décalage avec nos voisins. L'endettement des ménages et des entreprises rapporté au PIB est désormais le plus élevé des grands pays d'Europe. La dette publique est nécessaire, car elle permet le développement de nos services publics et soutient nos politiques sociales, culturelles, sanitaires, mais aussi économiques. Je rappelle que le Japon a une dette représentant 250 % de son PIB et ne voit cette réalité que comme un souci mineur, parce qu'elle est détenue en majorité par les Japonais. C'est l'économiste Bruno Tinel qui écrivait que,

Nous avons une proposition : il s'agirait d'orienter l'épargne des particuliers vers des obligations du Trésor grâce à une rémunération avantageuse et une défiscalisation, dès lors qu'elles seraient gardées sur le long terme. Sur la dette publique toujours, de nombreux économistes, et pas des moindres, s'accordent sur l'effacement d'une partie de notre dette détenue par la BCE et les banques. On évalue cette éventualité à environ 400 milliards d'euros, soit 17 % du PIB que l'État pourrait d'emblée injecter dans l'économie et qui permettrait surtout de prendre rapidement la bifurcation écologique et sociale sans laquelle les décennies à venir seront des périodes autrement plus dramatiques que ce que nous vivons. Nous pourrions aussi réfléchir à atténuer la charge de la dette par le pilotage maîtrisé d'une inflation douce. Derrière toutes ces propositions se cache un vrai enjeu, celui du maintien de notre souveraineté nationale : celle-ci ne doit plus être soumise aux aléas du marché. Garantir notre souveraineté, c'est aussi défendre notre économie au sens large, c'est défendre nos industries ; c'est défendre nos lieux de production ; c'est défendre nos produits ; c'est défendre nos emplois ; c'est défendre les territoires, et c'est ce qui nous permettrait d'être indépendants dans certains domaines majeurs comme les médicaments. Quoi qu'il en coûte », pour reprendre l'expression du Président de la République, nous devons repenser et dessiner une nouvelle politique industrielle. Le confinement a mis en lumière les enjeux liés à la relocalisation de la production, l'indispensable changement de nos manières de nous déplacer, de travailler, de consommer, mais surtout la nécessité d'une nouvelle stratégie industrielle et économique française. Quoi qu'il en coûte », nous devons soutenir par nos politiques sociales, nos concitoyens les plus précaires et les plus en difficulté. Pour un grand nombre de Français, ce confinement a aussi agi comme un révélateur des inégalités de logement et de la précarité de ceux qui exercent des métiers exposés au coronavirus et qui ont été nos premiers de tranchée. « Quoi qu'il en coûte », la transition énergétique doit se faire à marche forcée. Depuis trop longtemps, on court après la croissance pour rééquilibrer les comptes et diminuer le chômage de masse. pour quel résultat ? La dette publique et la dette privée explosent, et le chômage de masse ne disparaît pas. Il faut faire sans croire et sans souhaiter la décroissance, sauf une décroissance de l'empreinte écologique. Il nous faut cependant acter que nous sommes dans une économie en contraction, principalement à cause de la quantité d'énergie et de matières premières dont nous disposons qui s'amenuise ou que nous devons maîtriser. De cette manière, on peut concentrer le débat sur les stratégies à établir pour préparer un avenir commun, et non pour relancer le système tel qu'il était. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, il ne s'agit pas ici d'ergoter sur telle mission ou tel programme. Nous avons le devoir d'agir vite en répondant aux trois urgences aux trois urgences économique, sociale et écologique, parce que ce sont elles qui conditionnent notre avenir commun. Pour ce faire, nous devons nous extraire de nos croyances, des dogmes économiques que nous suivons que nous suivons depuis des décennies, pour construire un nouveau système économique, social et écologique en phase avec ce nouveau monde. Très bien

de passer en revue un certain nombre de conventions fiscales avec des pays étrangers qui, précisément, nuisent au contribuable national et au Trésor. Je conclurai en revenant

Le Gouvernement prend un gros pot de peinture verte et se met à verdir le budget, au lieu d'assurer la traçabilité des recettes à finalité environnementale, comme la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ou les redevances des agences de l'eau, qui sont censées financer des travaux évitant la pollution. Dans les deux cas, cela devient des recettes de poche du budget général.

Cela consiste à ne pas se disperser, à se fixer des priorités. Le Gouvernement semble avoir choisi une autre voie : « Nous nous occuperons de tout : des pistes cyclables, de l'isolation thermique des bâtiments, des énergies renouvelables, de l'artificialisation des sols ...

productivité globale ou compétitivité, progrès social et politiques environnementales ambitieuses peuvent aller de pair, mais [ ...] cela ne se fait pas spontanément. [Les politiques publiques] sont nécessaires, mais elles doivent être aussi bien conçues, cohérentes et privilégiant l'incitation sur la norme rigide ; s'attachant absolument à réduire " l'incertitude régulatoire ", génératrice de primes de risque élevées pour les investisseurs.

La méthode de mise en oeuvre nous intéresse également. Le Premier ministre, je le cite de nouveau, a indiqué que si de « grands débats » en matière d'écologie sont nécessaires, il souhaite davantage aborder le sujet depuis le terrain. Il a promis

Le Haut Conseil des finances publiques aura l'occasion d'actualiser ses prévisions au mois de septembre. Nous en tiendrons évidemment compte pour ce qui concerne l'équilibre du projet de loi de finances que nous présenterons.

des finances publiques. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire. M. le président du Sénat prendra acte de la clôture de cette session lorsque nous aurons reçu le décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. Cette information sera publiée au et sur le site internet de notre assemblée. Sauf élément nouveau, le Sénat se réunira le jeudi 1 octobre 2020, à 15 heures, avec l'ordre du jour suivant -Installation du bureau d'âge ; -Ouverture de la session ordinaire 2020-2021 ; -Allocution du président d'âge ; -Scrutin secret à la tribune pour l'élection du président du Sénat

Merci